de préserver les preuves et à la difficulté d'identifier l'agresseur, compte tenu du temps écoulé entre l'acte et la date à laquelle la justice s'en saisit. C'est pourquoi le prolongement à trente ans de la prescription prenant effet à compter de la majorité de la victime me paraît une Parce que ces délits ne doivent pas rester

Monsieur le président,

et même si on peut trouver des raisons particulières de rendre le viol subi par comme l'a rappelé

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin est ouvert.

de la proposition de loi relative à l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs. La séance est suspendue. ferait